Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,

ma part qu'il est de ces débats particulièrement utiles, même si nous ne sommes pas très nombreux ce soir. La qualité pallie la quantité En 1936, un projet de loi défendu par Jean Zay prévoyait la création d'une nouvelle école nationale d'administration,

à recruter ses principaux serviteurs dans une classe privilégiée restreinte dont les intérêts et les sentiments peuvent ne pas coïncider avec ceux de l'ensemble de la nation ».

de ses modalités sur la conduite de la politique de la Nation. Cette question n'a d'ailleurs cessé de jalonner les débats parlementaires, y compris sous la III République. Dès le début du XX siècle, alors que le recrutement par concours s'impose progressivement, on s'interroge sur la possibilité d'en finir une bonne fois pour toutes avec l'impression de cooptation que donnaient certaines pratiques de recrutement opaques. Il s'agit de doter la République d'un système de recrutement sur concours, sanctionnant uniquement le mérite du candidat, en rupture avec les réseaux de recrutement hérités des précédents régimes et du Second Empire. À la Libération, l'ENA est créée sous l'impulsion de Michel Debré. Elle a depuis formé nombre de personnalités éminentes de la République,

il est assez déstabilisant de remarquer que plusieurs des critiques de l'ancien régime de recrutement des hauts fonctionnaires demeurent malheureusement d'actualité. Les critiques ont surgi très tôt puisque, dès 1967, Jacques Mandrin- alias Jean-Pierre Chevènement,

Le pays avait eu, il y a trente ans, le cauchemar de la Synarchie, mais elle n'existait pas. Il découvre l'Énarchie, elle existe bel et bien. Il en ressent l'effroi d'un honnête homme qui se réveille ficelé par des brigands. » Nous reconnaissons là le tempérament de notre ancien collègue Jean-Pierre Chevènement Mes chers collègues, vous le savez, il ne s'agit pas de faire un procès aux grandes écoles françaises, qui sont pour la plupart aussi prestigieuses que performantes dans la production de nos élites- je pense à l'École polytechnique ou à l'École normale supérieure, pour ne citer qu'elles.

pose un sérieux problème de légitimité et d'acceptation de la décision produite par notre administration. L'ENA jouit d'un quasi-monopole pour la formation des cadres supérieurs de la fonction publique étatique, mais ses élèves ne sont pas assez représentatifs de l'ensemble de la Nation. On estime ainsi que près de 28 % des membres des grands corps de l'État auraient au moins un parent énarque. Cela fait tout de même beaucoup Comme en attestent les rapports annuels consacrés aux concours de recrutement de l'école, les grandes écoles parisiennes y sont surreprésentées, au premier rang desquelles Sciences Po Paris. La reproduction sociale fonctionne ici à plein régime

La possibilité d'offrir aux titulaires d'un doctorat une voie d'accès au concours interne sur titre a finalement été abandonnée en mars 2013 sous l'effet d'un certain nombre de pressions. Il existe donc une lente éviction sociale et territoriale qui commence de plus en plus tôt, puisque les formations préparatoires plébiscitées par le jury de l'ENA recrutent majoritairement dans le bassin parisien, pour ne pas dire dans quelques arrondissements parisiens bien précis. Certains parents choisissent même leur logement en fonction de la proximité des lycées les plus prestigieux, Saint-Louis ou Henri-IV. La formation dispensée à l'ENA pose également un certain nombre de problèmes : elle fabrique trop de hauts fonctionnaires stéréotypés, sur la forme et sur le fond. Lors de leur arrivée sur le terrain, ces derniers éprouvent souvent, à tort ou à raison, un sentiment de distorsion et d'inadaptation de leur formation à la réalité de leurs tâches quotidiennes. Le pire, c'est quand eux-mêmes ne se rendent pas compte de cette distorsion. Les critiques énumérées par les anciens élèves

de l'enseignement qu'ils avaient reçu : " L'École de Guerre nous a trompés. " » La trop forte porosité entre la sphère publique et les sphères économique et financière est également problématique : c'est la question du « pantouflage Cette porosité est encouragée par les dispositions normatives actuelles, destinées à permettre une meilleure « respiration » de la haute fonction publique, dont les membres peuvent se mettre en disponibilité.

Il est regrettable que des dispositions néfastes à la démocratie représentative soient souvent instillées par la haute administration. Les hauts fonctionnaires veulent souvent diminuer le nombre de parlementaires, mais rarement les effectifs des directions ministérielles Actuellement, les règles concernant le contenu de l'engagement décennal et le remboursement éventuel des frais de scolarité font défaut. Qui en assure le contrôle ? L'engagement décennal doit-il être considéré comme ayant été respecté lorsqu'un énarque est engagé prématurément dans un cabinet ministériel, par une administration européenne ou internationale, ou s'il se réoriente vers une carrière universitaire ? Puisque de nombreux énarques sont également d'anciens élèves de l'École normale supérieure, l'ENS, ou de l'École polytechnique, comment est calculée, madame la ministre, la durée totale d'engagement attendue ? Enfin, dans quels délais ces remboursements sont-ils La haute fonction publique devrait se recentrer sur sa raison d'être : exécuter les décisions des élus de la Nation. Or on observe de plus en plus l'inverse

J'ai été frappé par le mépris affiché par certains présidents, certes, minoritaires, vis-à-vis de la représentation parlementaire. L'inflation constante des directions centrales des ministères, la multiplication des autorités, agences et hauts conseils est une autre conséquence du poids des membres de ces grands corps, pour lesquels il faut parfois inventer des distinctions afin d'assurer leur avancement. Enfin, et surtout, il en résulte une véritable « diarrhée réglementaire », au point qu'on a parfois le sentiment que la machine administrative a inventé le mouvement perpétuel. Il est clair que, plus que pour toute autre, la pérennité de cette école repose sur sa capacité à intégrer ces critiques et à se réformer. Nous considérons qu'une telle réforme doit porter à la fois sur le recrutement, la formation et le cursus professionnel du haut fonctionnaire énarque. Plusieurs pistes peuvent être explorées. En matière de recrutement, la possibilité d'aménager des passerelles avec le milieu universitaire pourrait être étudiée, car elle pourrait apporter un peu de diversité. La refondation La refondation des épreuves pourrait être approfondie en veillant à évaluer la capacité des candidats à répondre à une commande politique et en accordant moins de poids à l'épreuve de culture générale.

: « Madame, pouvez-vous nous expliquer la différence entre pudeur, pudibonderie et pruderie ? » Ce moyen de sélection a atteint ses limites.

clarifier les règles de remboursement et fixer des délais précis. Il s'agit de s'assurer que la devise de l'École demeure « Servir sans s'asservir »-et non « se servir ». Le diplôme de l'ENA ne doit plus être considéré par quelques jeunes étudiants aussi brillants qu'ambitieux comme un ticket d'entrée dans une carrière politique accélérée, ou encore comme un moyen de parvenir au sommet de la direction d'une grande entreprise du CAC 40. Faire l'ENA, c'est d'abord être animé par le sens de l'État, c'est vouloir servir son pays en assistant le pouvoir politique, le seul qui bénéficie de la légitimité démocratique de l'élection, celle-là même qui lui permet de décider et d'assumer en responsabilité. Il s'agit donc, madame la ministre, non de supprimer l'ENA, mais de la réformer.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier mes collègues du groupe du RDSE et

qui, pour harmoniser et unifier les procédures de recrutement des différentes administrations, d'une part, et pour lutter contre le corporatisme inhérent à des cercles fermés, d'autre part, avaient eu l'idée de créer une procédure de recrutement et de formation unique. La démission pour l'un, le rejet du Sénat pour l'autre ont conduit au maintien d'un système dans lequel chaque corps s'organisait librement. Outre ces enjeux, se posait la question de la démocratisation de la haute fonction publique, sur la base d'une méritocratie républicaine et d'une égalité de fait entre classes dominantes et classes populaires. Au fond, c'était l'article VI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'il s'agissait de mettre en oeuvre. Par ailleurs, il faut aussi se rappeler le contexte de la création de l'ENA : notre pays était alors ravagé tant matériellement que moralement, notre administration

La création de l'ENA devait clairement permettre de faire émerger une nouvelle génération de hauts fonctionnaires, issus de tous les horizons, et pour qui les valeurs républicaines n'étaient pas juste un prétexte pour se dédouaner. Cette mission, c'est Thorez et Debré qui l'acteront, mais c'est tout le Conseil national de la Résistance qui l'initiera. La seconde question qui est posée est celle de l'accomplissement de cette mission par l'ENA aujourd'hui. À la réponse est forcément négative, et ce pour plusieurs raisons. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, dès les années soixante, avaient constaté que le projet émancipateur de l'ENA avait été biaisé et ne servait finalement qu'à la perpétuation des élites. Plus qu'une catégorie ou une classe, le monde de l'énarchie est devenu une caste se perpétuant de génération en génération. Ainsi, les « camarades de classe à l'école » deviennent « copains de promo à l'ENA

s'appuyer sur une école républicaine égalitaire, l'institution scolaire devant gommer les inégalités de capitaux au lieu de les creuser. Or, comme le rappelait le Conseil national d'évaluation du système scolaire en septembre dernier, la France reste la championne des inégalités à l'école parmi les pays de l'OCDE.

se limite peu ou prou à deux écoles elles-mêmes particulièrement élitistes, Polytechnique et Sciences Po. Même si cette dernière a, par le biais des conventions d'éducation prioritaire, tenté d'ouvrir plus largement ses portes, pas moins que le nombre de boursiers du 27 rue Saint-Guillaume n'atteint pas le tiers des élèves et que 65 % des étudiants sont issus des catégories socioprofessionnelles les plus élevées. Ces derniers représentent 82 % des nouvelles entrées à l'ENA s'est aggravée du fait de la suppression, en 1990, de la troisième voie, ouverte aux dirigeants associatifs et syndicaux, créée par Anicet Le Pors en 1983. Il s'agissait pour ce dernier de créer ce qu'il appelle « l'élitisme de masse ».

du projet d'Anicet Le Pors était la promotion aux plus hauts niveaux de l'administration de citoyennes et de citoyens de qualité, ayant fait la preuve de leur attachement au service public

La situation de l'ENA aujourd'hui, mélange d'homogénéité et de reproduction sociale, a des conséquences qui, en définitive, rejaillissent sur l'ensemble de l'administration et sur l'État. Tout d'abord, comme le montre Luc Rouban dans son étude sur les profils et trajectoires des énarques, les lignes entre le politique et l'administratif se sont brouillées depuis le début des années quatre-vingt. Il y a plusieurs raisons à cela, plutôt logiques d'ailleurs. D'une part, il ne faut pas oublier qu'une partie des énarques se sont lancés en parallèle en politique. De fait, leur pouvoir de nomination leur a permis de s'appuyer sur des gens de confiance pour mener leur action. Et qui d'autre que les fameux « copains de promo » pour le faire ? D'autre part, la technocratisation progressive de la politique a permis dans bon nombre de cas le renforcement de liens sur des fondements techniques et non idéologiques. Cette logique pouvait s'entendre

Qui peut dire aujourd'hui que les rapports d'éminents technocrates ne sont pas politiques ? Il est d'ailleurs à noter que les nouveaux énarques semblent souffrir des mêmes comme le relevaient les membres du jury d'admission à l'ENA en 2015 : « absence de sens critique », « incapacité de prise de hauteur » et « conformisme idéologique Et le profil des élèves admis à l'ENA, qui ont plutôt fait des écoles de commerce que des études de droit, ne peut qu'aggraver le problème. On se retrouve bien souvent avec des hauts fonctionnaires ayant un profil de gestionnaires privés bien plus que de cadres attachés au service public.

ait censuré le transfert à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du contrôle des départs vers le secteur privé des très hauts fonctionnaires et membres de cabinet. C'est en effet aujourd'hui une constante : les dix ans d'engagement au service de l'État et de l'intérêt général exigés des énarques en contrepartie de la gratuité de la formation ne sont que rarement À titre d'exemple, Bruno Bézard, mais il est loin d'être le seul, a quitté la direction générale du Trésor pour rejoindre un fonds d'investissement franco-chinois, Cathay Capital.

Reproduction des élites et homogénéité idéologique ont donc conduit à l'appauvrissement de la haute fonction publique, et donc des serviteurs de l'intérêt général, d'une part, et à des pratiques particulièrement douteuses de copinage entre les membres de cette caste,

madame la ministre, mes chers collègues, comme l'écrivait Marc Bloch, dont la loyauté à la République est indiscutable : « À une monarchie, il faut du personnel monarchique. Une démocratie tombe en faiblesse, pour le plus grand mal des intérêts communs, si les hauts fonctionnaires formés à la mépriser [ ...] ne la servent qu'à contrecoeur ». Le sens de l'État est la première qualité du fonctionnaire. Dans une démocratie, le président Mézard l'évoquait, le sens de l'État implique de respecter le principe démocratique et de se mettre au service du pouvoir élu. Malheureusement, cette qualité est l'une des plus difficiles à déceler au moment d'un concours. Elle ne se révèle en réalité qu'au cours d'une carrière, au travers des choix individuels du fonctionnaire, et se mesure à l'aune de sa propension à faire primer le bon fonctionnement de son service et de l'administration sur son destin personnel. On peut toutefois considérer que le fonctionnement actuel de l'ENA et le statut spécifique de la catégorie A+ présentent des défauts susceptibles d'affaiblir le sens de l'État de certains anciens élèves de cette école, comme celui des fonctionnaires d'autres catégories. Dans la continuité des constatations faites par Jacques Mézard, j'évoquerai la question des modalités d'affectation des énarques dans les différents corps, puis les difficultés managériales liées à l'imperméabilité de ces corps. En premier lieu, l'opacité qui entoure l'affectation de sortie des énarques dans les différents corps de l'administration est un facteur initial de frustration. Actuellement, tous les candidats d'une même voie- interne, externe, troisième voie -sont soumis aux mêmes épreuves, ce qui permet de recruter de bons généralistes. Chaque élève reçoit la même formation, malgré la différence des postes accessibles à la sortie de l'école : conseiller de tribunal administratif, administrateur civil au ministère de l'agriculture, conseiller des affaires étrangères ou inspecteur général de l'administration ... La cérémonie de l'« amphi-garnison qui clôture la scolarité à l'école, au cours de laquelle les élèves choisissent leur affectation successivement en fonction de leur rang de sortie, ne permet pas d'aiguiller les élèves vers les carrières les plus adaptées à leurs compétences. Un individu ayant une formation d'économiste pourra ainsi être nommé au Conseil d'État. Surtout, la performance de l'élève au cours de ses deux années d'école et son classement final auront un impact très fort

On pourrait pourtant imaginer différentes solutions : les candidats pourraient choisir une épreuve majeure en fonction du corps qu'ils souhaitent intégrer lors du concours d'entrée ou l'affectation par classement pourrait se faire dès l'entrée à l'École, sur la base des notes obtenues au concours. La formation des élèves pourrait ainsi être calibrée en fonction de leur future affectation. Saluons néanmoins l'ouverture accrue de l'École aux entreprises. Cela étant dit, peut-être ne serait-il pas inutile que les futurs administrateurs civils et magistrats puissent effectuer un stage au sein du Parlement En second lieu, l'existence d'une catégorie A+ implicite et rigide cause de nombreuses difficultés managériales. Tout d'abord, cette catégorie s'est imposée hors de tout cadre législatif, puisque la loi du 11 janvier 1984 1984 ne prévoit que trois catégories distinctes : A, B et C. Elle a seulement été définie dans le rapport annuel 2009-2010 de la DGAFP. Il s'agit d'un frein considérable à la promotion de la performance au sein de la fonction publique, puisque, à travail égal ou supérieur, un cadre de catégorie A ne pourra jamais parvenir à un niveau d'intéressement égal à celui d'un cadre de catégorie A+, sauf à repasser des concours internes. Pourtant, en raison du maintien de concours d'accès parallèles pour des fonctions nécessitant une certaine spécialisation, on constate l'existence de différences de traitement substantielles entre un énarque et un autre fonctionnaire à des postes similaires. C'est notamment le cas au ministère des affaires étrangères, dans les tribunaux administratifs et les chambres régionales des comptes. Un alignement des grilles de traitement doit être envisagé, dans un souci d'équité. De façon plus ambitieuse enfin, la différenciation de la catégorie A et de la catégorie A+ pourrait être repensée. Il faudrait dynamiser les outils de promotion interne qui doivent être fondés non seulement sur l'expérience, mais aussi sur la performance. Il faut approfondir le travail accompli dans ce sens depuis la remise du rapport Diefenbacher. Ainsi, l'existence même de l'accès direct aux grands corps pourrait être remise en cause en s'inspirant du fonctionnement de l'ordre judiciaire. Il serait peut-être bon de réserver en partie l'accès au Conseil d'État, à la Cour des comptes et à l'Inspection générale des finances aux fonctionnaires ayant fait preuve de leurs mérites dans le long terme, et non pas seulement lors du concours initial. En conclusion, cette refondation doit être conçue en parallèle d'une réflexion sur la lutte contre le pantouflage. La création de commissions de déontologie ne semble pas suffisante. Vous l'aurez compris, il s'agit dans tous les cas de valoriser la carrière des hauts fonctionnaires démontrant sur le long terme leur sens de l'État,

et dont beaucoup de parents, souvent issus eux-mêmes de la fonction publique, rêvent pour leurs enfants, parce qu'elle est dans leur esprit synonyme de réussite. Il suffit, en effet, de se pencher sur le parcours de certains des responsables politiques ou cadres supérieurs de diverses entreprises en vue pour constater que l'ENA fait l'ENA fait partie des écoles dont sont issus, depuis la fin de la guerre, un certain nombre de dirigeants de notre pays. À l'inverse- et c'est sans doute la contrepartie des rêves que l'ENA a pu susciter dans certaines familles ou certains milieux

déception de ne pas avoir réussi le concours, regret de ne pas être sorti avec un classement permettant d'accéder directement à un grand corps, sentiment que les candidats issus de certains milieux socioprofessionnels ont plus de chances que d'autres d'y accéder, etc. Il y a toujours une bonne excuse à faire valoir. Comme disait ma grand-mère : « il vaut mieux faire envie que pitié ». Il est donc tout à fait naturel que cette école, que cette école, dont beaucoup de parents rêvent pour leurs enfants, fasse l'objet d'autant de critiques que de louanges. Faut-il pour autant supprimer l'ENA ? Si oui, par quoi la remplacer ?

Quels sont donc les reproches que l'on entend le plus souvent ? D'abord, celui de ne plus jouer le même rôle de démocratisation de l'accès à la haute fonction publique qu'à ses débuts. Alors qu'avant 1945 chaque filière de la fonction publique organisait son propre recrutement et avait naturellement tendance à puiser dans le même milieu socioprofessionnel de génération en génération, force est de constater que la création

Il n'y a pas que des fils de préfets ou de conseillers d'État qui entrent à l'ENA, et je crois pouvoir dire que j'en suis un des nombreux exemples, moi qui suis le fils d'un couple de petits agriculteurs n'ayant chacun que leur certificat d'études. J'étais d'ailleurs le seul fils d'agriculteur dans ma promotion. Peut-être était-ce un alibi pour l'ENA ? Je n'en sais rien. Alors oui, si la création de l'ENA a constitué une sorte de rempart au népotisme et, de manière générale, à la politisation de de l'administration publique qui existait à l'époque, force est cependant de constater un paradoxe, celui de la faible diversification de son recrutement. Si l'on se réfère à une étude menée par deux chercheurs

de chaque promotion de l'ENA, suivis par 12 % d'élèves issus de la catégorie des professions intermédiaires, 9 % de familles d'agriculteurs ou artisans, et seulement 6 de familles d'employés et d'ouvriers. Il faut aussi constater que l'on observe peu ou prou les mêmes répartitions d'origines socioprofessionnelles à Sciences Po, à l'École normale supérieure ou à l'École polytechnique.

Alors, quelle solution face à cette sorte de « reproduction des élites » ? J'avoue ne pas avoir la réponse. Un autre reproche est souvent adressé aux énarques, celui de peupler les cabinets ministériels et d'avoir une forte- certains diraient trop forte -influence sur les politiques qui sont menées par les divers gouvernements dans certains domaines, quelle que soit leur couleur politique. Il est vrai l'on fait parfois le même reproche à certains professionnels de l'éducation nationale s'agissant de la politique scolaire. Nul n'ignore que le ministère de l'éducation nationale est truffé d'enseignants et que, s'il est

On touche là directement, je crois, à la responsabilité du politique. Suffit-il de remplacer un énarque par un autre dans un cabinet ou de remplacer un énarque par un non-énarque pour mieux régler ou régler différemment un problème ? Ce serait tellement simple si cela suffisait ! Et cela se saurait ... En tout état de cause, s'il est clair qu'un membre du Gouvernement est d'abord un politique, il est non moins clair qu'il a besoin de travailler avec des collaborateurs connaissant les rouages de l'administration. Et force est de reconnaître que, dans certains ministères, ce sont souvent des énarques qui occupent des postes à responsabilités parce que, précisément, les administrateurs issus de cette école sont ceux qui connaissent le mieux le fonctionnement interne et les moyens dont dispose l'État. Dans certains ministères, les postes à responsabilités sont tenus par des magistrats ou des membres de l'éducation nationale, pour ne citer que ces deux exemples. Même problème, même solution ! Ces ministères sont-ils mieux gérés que ceux qui sont peuplés d'énarques et les politiques qu'ils mènent sont-elles plus efficaces ? Je ne me permettrai pas de répondre ni de dire ce que j'en pense. Alors, quelles solutions, si l'on considère que l'ENA pose problème pour notre pays ? Supprimer cette école n'arrangerait rien. Nous avons besoin d'une haute fonction publique formée et préparée aux responsabilités. peut toutefois penser à des améliorations, comme le fait de rendre plus professionnel et moins théorique l'accès au concours de l'ENA à partir d'un certain niveau de responsabilités et de donner peut-être une plus grande part,

ou décentralisées, dans des entreprises, des collectivités ou autres structures, dont les élèves seront éventuellement appelés ultérieurement à réglementer ou à superviser les activités Peut-être aussi faut-il que les politiques fassent preuve d'une plus grande implication dans la préparation et la mise en oeuvre des décisions relevant de leurs ministères

Faisons-nous bien notre travail si nous votons, dans une loi, une décision de principe et si nous ne regardons pas la manière dont les administrations centrales la mettent en oeuvre ? mettent en oeuvre ? Là aussi, il y a quelque chose à faire sans qu'il soit nécessairement besoin de taper sur l'ENA. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire, sans doute trop longuement, à propos de l'ENA, en osant, pour conclure, parce que le problème n'est pas simple à régler, paraphraser Churchill : l'ENA est pour l'administration publique la pire des formations, à l'exception de toutes les autres.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, une scolarité déconnectée de la réalité, l'inadaptation du contenu des enseignements aux nouveaux enjeux du monde contemporain, l'obsession du classement, la responsabilité des élites dans la défiance envers les institutions politiques et administratives, les griefs formulés ici même à l'encontre de l'École nationale d'administration sont nombreux et nous interrogent. Je remercie donc très vivement le groupe du RDSE et son président, Jacques Mézard, d'avoir fait inscrire à notre ordre du jour ce débat sur la nécessité de supprimer ou non l'ENA. Si la manière dont sont recrutés et formés les hauts fonctionnaires, et plus généralement même l'existence des grands corps de l'État, ne nous donne pas satisfaction, ces questions doivent être réglées. Le recrutement des énarques pose la question de savoir qui sont nos élites. Le constat est édifiant, cela a été dit par tous les orateurs : ces dernières sont majoritairement masculines, alors que les filles réussissent plutôt mieux à l'école, issues des mêmes milieux sociaux et des mêmes écoles. Cette absence totale de diversité n'est absolument pas en adéquation avec les besoins de notre société :

Le système actuel comprend tout de même des moyens de diversifier la haute fonction publique, avec le troisième concours s'adressant aux actifs du secteur privé, aux élus et aux responsables associatifs.

Développer la diversification, cela passe aussi par l'éducation pour lutter contre l'autocensure, évoquée par la présidente Assassi, qui explique aussi que les jeunes issus de milieux modestes ou les femmes tentent moins d'entrer

L'évolution de notre haute fonction publique passe également par la formation initiale et continue des énarques. Le mouvement enclenché en 2016 est encourageant : il était temps ! Des changements importants ont été engagés depuis

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais d'abord rendre hommage aux très nombreux anciens élèves de l'École nationale d'administration que j'ai pu rencontrer dans des préfectures, des ministères, des établissements publics et qui m'ont souvent frappé par leur haut sens de l'intérêt public et du service public. Il y a tellement de « marronniers », comme l'a dit Jacques Mézard, consistant à imputer à cette école quelques-uns des maux de la société qu'il faut aussi rendre hommage à ceux qui ont créé cette école,

Je ne voudrais pas que l'on fasse finalement une erreur de raisonnement, qui serait sanctionnée dans beaucoup de concours, consistant à créer des rapports de causes à effets sans jamais les prouver.

? Certes, il existe un antiparlementarisme dans notre pays, mais je ne crois pas qu'on puisse l'imputer aux énarques plus qu'à d'autres. D'ailleurs, au sein du Parlement,

d'un itinéraire relevant de la méritocratie républicaine ; il ne faut pas le dénigrer. La vérité, c'est que la démocratisation de l'enseignement est sans doute, dans certains de ses aspects, en régression. Les chiffres que l'on donne quant à l'origine sociale des élèves valent pour l'ENA aussi bien que pour l'École polytechnique, HEC et beaucoup de grandes écoles de ce pays.

mais, si l'on veut régler cette question, il faut beaucoup de temps scolaire, se concentrer sur les savoirs fondamentaux dès l'école,

loin. Notre école est à refonder autour de l'idée d'une école de l'exigence. Cela a été réalisé dans l'histoire, à une époque où beaucoup moins de jeunes faisaient des études jusqu'au baccalauréat. je crois que la source du problème est beaucoup plus profonde, elle se trouve dans l'ensemble de notre conception de l'enseignement dès le départ.

être admis dans des classes préparatoires aux grandes écoles où exercent d'excellents enseignants qui ne sont pas tenus à des activités de recherche

à analyser est primordial, et je ne suis pas forcément convaincu par les discours qui, à l'école élémentaire comme à l'ENA, vantent une grande dispersion des séquences de formation. On veut ouvrir l'école sur tout c'est très bien, mais il faut d'abord assurer le fondamental. Je dirai la même chose pour l'École nationale d'administration. Les stages, que ce soit dans une administration ou une collectivité locale, locale, dans une ambassade à l'étranger ou dans une entreprise, sont très précieux et bénéfiques, mais il faut aussi que le reste de la formation soit substantiel.

administrateurs de nombreux ministères, et même du Sénat ou de l'Assemblée nationale, ne manquent pas de faire des cours à l'ENA, et ils le font très bien. Mais ne faudrait-il pas réfléchir à une structure permanente plus forte, avec une pédagogie et des programmes mieux définis ? Le fait de disposer de programmes mieux définis n'est pas antinomique du fait de donner à l'enseignement le caractère général qui me paraît nécessaire, étant entendu, bien sûr, qu'un enseignement général qui n'a pas d'ouverture sur les réalités professionnelles est un enseignement à la généralité duquel il manque quelque chose. Enfin,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans les prochains mois, trois élections majeures se succéderont : deux élections parlementaires et une élection présidentielle. Comme à chaque grand renouvellement, nous assisterons à la valse des cabinets ministériels, qui verra des énarques, directeurs de cabinet ou conseillers, être remplacés par d'autres, avec le même profil. Dans le reste du système, des directeurs d'administration centrale changeront, des préfets, des ambassadeurs. Tous, ou presque, seront remplacés par le même modèle. Corps de direction des administrations, corps préfectoral, corps diplomatique, corps des magistrats, corps d'inspection générale ... et combien de ministres et de parlementaires : tous sont passés sur les bancs de l'École nationale d'administration. C'est vrai, les énarques sont partout, car ils sont formés pour le service de l'État au plus haut niveau. Leur concours est difficile, leur formation rigoureuse. L'école demeure prestigieuse en France et constitue toujours un modèle à l'étranger- du moins, nous l'espérons Tout semble normal, voire excellent. Pourtant, la défiance vis-à-vis de l'ENA et des hauts fonctionnaires qu'elle forme ne fait qu'augmenter. De tous les bords politiques, les « modernistes », en tout cas ceux qui se revendiquent comme tels, proposent de réformer, voire de supprimer l'ENA. La plupart du temps, ils en sont eux-mêmes issus et ne l'ont critiquée qu'après avoir tiré profit du statut de haut fonctionnaire et du réseau des anciens élèves. Un ancien ministre du redressement productif tirait encore récemment à boulets rouges sur l'école, avant que la presse ne lui rappelle l'influence qu'il avait laissée aux énarques de son cabinet, lui qui avait raté le concours Supprimer l'ENA ? La réponse la plus tentante serait de répondre par l'affirmative, car cette école n'a pas toujours bonne presse dans l'opinion publique. Mais est-ce vraiment elle qui exaspère ou l'attitude de certains de ceux qui en sortent ? Est-ce le statut protecteur de la fonction publique, le pantouflage ou le poids excessif des grands corps qui irrite ? Sans doute les causes du désamour sont-elles multiples. Il est vrai que, de cadre de formation des grands serviteurs de l'État, l'ENA est devenue l'antichambre du pouvoir. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas favorable à la confusion des genres, et c'est pourquoi une claire séparation entre élus et hauts fonctionnaires me semble nécessaire. Les énarques devraient démissionner de leurs fonctions pour faire de la politique. La politique, c'est une vocation et un risque, et non pas une ligne à ajouter à son CV Mes chers collègues, avec la fin du cumul des mandats cette année, il existe bien un danger de voir les élus de terrain progressivement remplacés par des apparatchiks ou des hauts fonctionnaires, catégories moins exposées que les autres. De plus, la vocation du service public n'est plus ce qu'elle était. Ainsi, en cinquante ans, on est passé du cadre supérieur au service de l'État, finissant chef de service, au dirigeant « multicarte » migrant d'un service à un cabinet, puis à un établissement public, pour aller en entreprise et revenir, avant de repartir pour finir comme président d'une banque d'affaires. Par ailleurs, je regrette le manque relatif de culture européenne des élèves, bien que leur établissement fût symboliquement déplacé à Strasbourg et leurs cours sur l'Union renforcés. J'aimerais ainsi que davantage de ces jeunes gens, avec leur niveau d'études, se présentent prioritairement aux concours